Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d'accueil sur le territoire français.

pour les préjudices subis par les harkis et leurs familles à leur arrivée en France. L'indignité des conditions de vie et d'accueil des harkis, notamment dans les camps et les hameaux, ainsi que les privations de liberté, a entraîné des souffrances et des traumatismes pour des milliers de femmes et d'hommes. La reconnaissance de la responsabilité prend la forme d'une indemnisation forfaitaire symbolique. Nous considérons que les critères proposés par ce texte sont trop restrictifs pour permettre une indemnisation de l'ensemble des harkis. En ne retenant que les personnes ayant séjourné dans les camps de transit et les hameaux- et encore, pas tous ! -, ils excluent de fait plusieurs milliers de harkis qui sont arrivés par leurs propres moyens ou qui ont séjourné dans d'autres lieux. Ensuite, le critère de durée de séjour dans une structure n'est pas satisfaisant. En créant une distinction selon les personnes qui ont résidé moins de quatre-vingt-dix jours dans un camp, le Gouvernement divise inutilement les familles de harkis. Surtout, ce critère ne prend pas en considération les circonstances et préjudices particuliers et personnels, par exemple le décès survenu dans un camp. C'est toute la limite d'une indemnisation forfaitaire. Ensuite, nous regrettons le choix de la date limite pour bénéficier de l'indemnisation, à savoir le 31 décembre 1975, alors que les structures ont continué d'accueillir des familles de harkis. Pour l'ensemble de ces raisons, nous nous abstiendrons sur cet article 2. La parole est à M.

madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, cet article 2 constitue, avec l'article 1, le point crucial de ce projet de loi, puisqu'il porte sur les mesures de réparation. Comme l'ensemble de ce projet de loi, cet article 2 n'est pas à la hauteur du drame que les harkis ont vécu. Je voterai donc contre. Premier point sur lequel je suis en désaccord, l'indemnisation ne repose que sur la durée de séjour dans les structures destinées à accueillir les harkis.

Leur seul tort est de ne pas avoir vécu entourés de barbelés ... En commission, j'ai tenté d'ouvrir cette indemnisation à tous, mais, bien évidemment, le couperet de la recevabilité financière Second point sur lequel je suis en désaccord, cette indemnisation ne prend pas en compte le fait que nombre de harkis de la première génération ayant vécu ce drame ne seront jamais indemnisés,

à son conjoint ou à sa conjointe, ou bien, à défaut, à ses enfants. Troisième point sur lequel je suis en désaccord, il s'agit ici d'une réparation sur la base d'une somme forfaitaire et d'un barème froid,

Poumirol, sur l'article. Nos collègues l'ont rappelé, cet article crée un mécanisme de réparation lié à l'engagement de la responsabilité de l'État et en fixe les principales modalités.

Par conséquent, conditionner ce droit à réparation au passage dans une structure déterminée rompt avec le principe constitutionnel d'égalité des citoyens. Il est important que tous les harkis et leurs familles puissent être entendus et présenter une demande individuelle de réparation du fait du préjudice qu'ils ont subi.

de loi d'obtenir réparation « en tant que victimes d'une politique de ségrégation sociale ». En effet, la ségrégation se définit comme une « action par laquelle on met un élément à part, on le sépare de l'ensemble

sur le territoire métropolitain, constitue, de fait, une forme de ségrégation sociale. L'ambition de ce projet de loi étant de reconnaître la responsabilité de la France du fait des conditions indignes de l'accueil des personnes anciennement de statut civil de droit local et de leurs familles, rapatriées d'Algérie,

il ne semble pas opportun d'apporter une telle précision, qui, du reste, n'aurait aucune incidence sur l'accès au droit à réparation. Celle-ci consacrerait en effet dans la loi un terme particulièrement fort, qui signifie la séparation des personnes pour l'accès au logement, à l'éducation, aux soins, à l'emploi ou aux transports. La commission demande donc le retrait de cet amendement,

de la liste des structures concernées par le mécanisme de réparation. L'objet de l'amendement est donc en partie satisfait, car cette commission aura un pouvoir de proposition relativement

des allocations déjà perçues. Ces allocations, je le rappelle, étaient fondées sur le principe de la solidarité sociale et non sur une compensation liée au comportement défaillant de l'État, ce qui est l'objet du présent Aussi, selon nous, il est important d'exclure clairement du calcul desdites allocations les montants déjà perçus. Qu'il n'y ait pas de fongibilité entre les deux nous paraît primordial, et il convient que cela soit inscrit clairement dans la loi.

L'article 2 est très clair concernant les sommes pouvant être déduites du montant de la réparation. Aucune des autres aides et allocations diverses versées aux anciens supplétifs et aux membres de leurs familles n'étant accordée à titre de réparation de ce préjudice, il ne paraît pas nécessaire d'apporter la précision proposée. L'amendement étant satisfait,

que ce soit sur le sol algérien ou sur le territoire français. Nous pourrons ainsi mener des auditions d'historiens, de chercheurs, d'universitaires et de descendants de harkis pour être au plus près de la vérité historique. Nous suivrons également les travaux de la commission indépendante instituée par l'ONACVG. Il est aussi dans les missions du Parlement que d'engager un travail de fond avec le Gouvernement. À l'issue de cette mission d'information, un rapport sera rendu public au plus tard le 31 décembre 2022. Quel L'initiative des travaux de contrôle des parlementaires relève de la conférence des présidents de chaque assemblée, des commissions permanentes et des groupes parlementaires, qui disposent d'un « droit de tirage » annuel. Elle ne relève en aucun de la loi.

Je veux saluer, tout d'abord, le travail qui a déjà été effectué par l'ONACVG sur cette question. Ainsi, en 2014, le plan harkis prévoyait le lancement d'une campagne de recueil de témoignages oraux de harkis, afin de collecter et de garder la trace des expériences vécues. Ces témoignages sont mis à disposition du public, mais aussi des chercheurs, dans le cadre de leurs travaux sur la mémoire des harkis. Néanmoins, une difficulté subsiste quant au recueil de ces témoignages : la barrière de la langue. Il faudra donc veiller à ce que des traducteurs soient présents. Le deuxième problème est la valorisation de ces mémoires et de ces archives. Il faut soutenir toutes les actions qui y participent. Pour cela, l'ONACVG a conclu des partenariats avec certains services départementaux d'archives, afin d'organiser des journées d'études sur l'histoire et la mémoire des harkis. J'insiste également sur l'importance de la transmission de cette histoire des harkis. Il est essentiel qu'elle puisse être enseignée, en particulier dans les établissements scolaires. Le ministère de l'éducation nationale doit s'impliquer pour assurer une diffusion large et pérenne de la connaissance sur ce sujet. À titre d'exemple, des interventions réunissant « quatre voix »- un ancien supplétif, un ancien partisan du FLN, un ancien appelé et un rapatrié d'origine européenne -ont été organisées dans certains établissements. Ces expériences Ces expériences sont à mon sens très importantes pour permettre la transmission des différentes mémoires de la guerre d'Algérie, ainsi que leur apaisement. Il faut que l'histoire de France, même la plus douloureuse, soit connue et reconnue par l'ensemble de nos concitoyens. C'est une condition du vivre-ensemble. La parole

dans l'histoire. La mémoire est passagère, puisqu'elle s'en va avec les êtres humains qui meurent, et elle est fragile. Il faudrait donc, parallèlement à la mémoire, qu'une qu'une place plus grande soit accordée dans les livres d'histoire aux recherches

Conformément à ce changement de rattachement administratif, il tend également à modifier le II de l'article 3, afin de préciser que les représentants de l'État siégeant au sein de cette commission seront désignés par le Premier ministre, et non plus par le ministre chargé des anciens combattants. De plus, en complément de ce nouveau positionnement de la commission, le présent amendement tend à conforter l'ONACVG dans sa mission d'instruction des demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 2 du projet de loi et à prévoir que l'établissement public assurera des missions de soutien nécessaires au bon fonctionnement de la commission.

et une aide à la décision. Une telle mesure permet ainsi de compléter les modifications apportées par la commission des affaires sociales, qui a souhaité renforcer l'indépendance de cette commission.

L'amendement n°

Enfin, elle aura la faculté de proposer des évolutions de la liste des lieux dans lesquels il est nécessaire d'avoir séjourné pour bénéficier du mécanisme de réparation. Cet amendement vise à compléter ces missions, en prévoyant spécifiquement un accès prioritaire à la commission pour les anciens combattants harkis et moghaznis et pour le personnel de diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilé, et cela peu importe leurs conditions de rapatriement et d'accueil sur le territoire national. En l'état actuel du texte, une telle compétence n'est pas encore prévue. Cet amendement vise à combler ce manque. Je suis certain, mes chers collègues, que vous serez tous naturellement sensibles à cette écoute accordée aux harkis combattants. Ainsi la commission sera-t-elle compétente pour entendre, à leur demande, ces anciens combattants. Elle pourra leur proposer, au regard de la situation individuelle des personnes entendues, toute mesure de reconnaissance appropriée compte tenu des services qu'ils ont rendus à la Nation. Je remercie mes collègues des nombreux groupes qui ont cosigné cet amendement et qui le soutiennent, parce qu'ils sont convaincus de sa portée.

Vous ne prévoyez donc pas une véritable ouverture à l'indemnisation. Pour toutes ces raisons, je suis contre ces amendements identiques, dont le défaut est d'être plus restrictifs que l'amendement Retailleau que nous allons examiner.

Cet amendement a pour objet d'intégrer aux missions de la commission nationale indépendante la tâche de chiffrer le montant global des réparations, en fonction de l'évaluation des préjudices effectifs et sociaux subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de leurs familles, qu'il s'agisse des atteintes à leur dignité, des conditions de dénuement dans lesquelles ils ont été contraints de vivre, ou encore des préjudices sociaux tels que la privation d'activité professionnelle. L'objectif est également de ne pas fonder cette réparation uniquement sur le nombre de mois passés dans les lieux ciblés par la loi, mais de permettre à la commission de poursuivre une évaluation plus précise des préjudices et de travailler à une meilleure réparation en fonction des résultats de ses travaux. Le montant global des réparations doit en se fonder mathématiquement sur le nombre de mois passés dans des camps ou des hameaux de forestage, mais être déterminé sur le fondement de l'évaluation des préjudices subis par les harkis. Est aussi visée ici l'équité de traitement dans la réparation individuelle des préjudices subis, sans pour autant remettre en cause le dispositif actuel, mais davantage son chiffrage global, fixé de manière prédéterminée. Cette proposition est conforme et fidèle à une approche visant à la réalisation d'un véritable travail d'évaluation des préjudices subis par les harkis, seul à même de rendre justice de manière incontestable et incontestée,

Le système prévu par le projet de loi permet d'indemniser les intéressés, à la seule condition qu'ils apportent la preuve d'un séjour dans une structure fermée, établissant ainsi une présomption de préjudice. Le chiffrage proposé n'aurait donc pas de conséquence sur le mécanisme forfaitaire à l'article 2. Il est préférable,

associations. Elle ne remet absolument pas en cause la répartition des rôles entre la commission et l'ONACVG, lequel sera bien chargé d'assister la commission et d'exécuter ses décisions, comme le prévoit l'article 3. Les conditions d'indépendance de cette commission ont été renforcées dans le texte et son rattachement au Premier ministre,

n° 8 rectifié. Cet amendement vise à élargir la période de prise en compte de la commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis, afin que chacun puisse prétendre aux réparations sans que de dramatiques effets de seuil

soit utilisé, afin de participer à la connaissance de cette période de notre histoire. Ces fonds doivent être enseignés et rendus publics, afin de participer au nécessaire et fondamental travail de mémoire sur le long terme.

Néanmoins, cette mission relève du code du patrimoine et du service public d'archives compétent, qui mettra en oeuvre le contrôle scientifique et technique permettant de garantir la conservation et l'accessibilité dans les meilleures conditions

Je rappelle que le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif seront tous deux représentés dans cette commission, où siégeront notamment un membre du Conseil d'État, un magistrat de la Cour de cassation et des représentants de l'État désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants.

qu'il n'était pas souhaitable de multiplier la participation des sénateurs à des organismes extraparlementaires. En outre, les prérogatives des parlementaires en matière de contrôle et d'évaluation permettront de suivre et de contrôler les activités de cette commission de reconnaissance et de réparation. Si nous y siégeons, nous serions en quelque sorte

madame la ministre,

De même, la désignation des maires des communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées à l'article 2 du présent projet de loi interviendra en concertation avec les associations d'élus, Vous l'aurez compris, mes chers collègues, cet amendement a pour objet d'assurer l'indépendance des membres siégeant au sein de la commission, et d'associer pleinement les autorités concernées au processus de désignation. Quel est l'avis de la commission

L'amendement tend à préciser utilement les conditions de désignation des membres de la commission. Il vise à renforcer les garanties d'impartialité conférées par le projet de loi, en précisant que les maires des communes ayant accueilli sur leur sol

l'allocation de reconnaissance touche 4 787 harkis et veuves, l'allocation viagère 1 117 veuves, les compléments de bourses pour les enfants scolarisés 99 enfants. L'aide spécifique au conjoint survivant bénéficiait à 35 personnes en 2019. l'aide au rachat de trimestres de cotisations retraite pour des enfants de harkis n'a aucun bénéficiaire, en raison de conditions d'âge trop restrictives. Plutôt que de maintenir un empilement de dispositifs qui s'adressent à quelques centaines de familles, ce texte aurait pu accorder une indemnisation unique pour tous les harkis.

présenter l'amendement n° 65. Le présent amendement a pour objet d'allonger de quatre à six années la période au titre de laquelle les veuves des anciens membres des formations supplétives ou assimilés peuvent solliciter le bénéfice des arrérages de l'allocation viagère auxquelles elles auraient pu prétendre au titre des années

de plusieurs milliers d'euros la somme versée aux veuves de harkis décédés cinq ou six ans avant la date de leur demande de bénéfice de l'allocation viagère. Cet amendement tend également à étendre la faculté de solliciter ces arrérages aux futurs bénéficiaires de l'allocation viagère

arrêts dans l'objet de cet amendement. Par ailleurs, l'article 5 de la loi précitée ne détermine pas les éléments constitutifs de l'infraction et ne fait pas référence à la loi sur la presse. Or, en vertu du principe de légalité des peines, aucune peine ne peut être prononcée à raison d'un fait qui n'est qualifié par la loi ni de crime, ni de délit, ni de contravention.

après les accords d'Évian. Toutefois, cet article est lacunaire, puisqu'il n'institue aucune sanction pénale. Le présent amendement vise donc à remédier à cette lacune, en instaurant une sanction pénale au travers d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à douze mois.

les insultes faites aux harkis ne peuvent plus être acceptées, compte tenu du parcours et de l'histoire de ces derniers ; nous l'avons démontré tout au long de cette soirée. À plusieurs reprises, le législateur a tenté de réprimer ces actes, sans réel succès.

et la diffamation commises envers un harki en raison de sa qualité, ainsi que pour l'apologie des crimes commis contre les anciens supplétifs, après les accords d'Évian. La loi du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées assimile l'injure et la diffamation à l'encontre des forces supplétives à celles qui visent les forces armées, pour lesquelles les articles 30 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoient déjà des sanctions, à savoir 45 000 euros d'amende pour la diffamation et 12 000 euros pour l'injure. Elle permet également aux associations défendant les intérêts moraux et l'honneur des harkis et justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de se constituer partie civile. L'injure et la diffamation adressées à une personne considérée individuellement en raison de sa qualité réelle ou supposée d'ancien supplétif relèvent en revanche du droit commun. Les intéressés sont donc libres d'engager des poursuites pénales au titre de l'injure ou de la diffamation de droit commun. L'institution d'un régime pénal spécifique pour l'injure et la diffamation commises envers une personne à titre individuel du fait de sa qualité d'ancien supplétif pourrait se révéler contraire au principe d'égalité devant la loi et faire l'objet de la censure du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, une telle mesure ne manquerait pas de faire émerger des demandes comparables émanant d'autres communautés.

injures, propos négationnistes, incitations à la haine -que subissent nos compatriotes harkis.

Néanmoins, j'adhère à ce que viennent de dire nos collègues sur la question des insultes faites aux harkis et je pense que, au travers de ce texte portant « reconnaissance » et « réparation », nous nous honorerions en faisant en sorte que ces insultes ne soient plus possibles, ou, en tout cas, qu'elles soient réprimées.

Le fait que ces injures particulières puissent être réprimées de façon efficace constituera un signe fort de reconnaissance et de réparation.

Il s'agit d'évoquer, dans l'intitulé du projet de loi, les conditions de « vie », plutôt que les conditions de « séjour » dans les structures dédiées à l'accueil des anciens supplétifs et de leurs familles.

l'avis du Gouvernement ? L'article 2, qui définit les conditions de mise en oeuvre de la réparation, fait bien référence aux conditions de « séjour » dans ces mêmes structures.

par les personnes rapatriées ayant vécu dans des structures de transit et d'hébergement particulièrement indignes, avec privation de liberté et tutelle administrative.

leur abandon et la responsabilité de l'État dans les conditions indignes de leur rapatriement après les accords d'Évian, est un pas de plus vers une mémoire apaisée.

Nous veillerons aussi à ce que la mémoire des harkis continue de vivre et d'être transmise, notamment grâce au travail de l'ONACVG.

nos divergences, chacun de nous partage la même volonté de réparer cette faute de l'État au regard de l'indignité de l'accueil et du séjour des harkis et autres rapatriés d'Algérie et de leurs familles dans ces camps et hameaux de forestage, d'abord au nom de la justice, mais aussi au nom du nécessaire chemin vers la réconciliation nationale. J'ai regretté d'entendre que la seule la seule différence de traitement n'était liée qu'à l'existence de barbelés. Allez dire cela à ceux qui ont vécu des années dans ces structures, qui ont perdu des enfants en raison du froid et de la faim qui n'ont eu d'autre voie que d'accepter une tutelle administrative- après avoir fui, ils se sont retrouvés enfermés ! Il est de notre devoir de ne pas jeter de l'huile sur le feu et sur la douleur des harkis. Je me réjouis que nos travaux nous aient permis d'avancer un peu plus sur la commission nationale de réparation et de conciliation, en sécurisant son indépendance et en élargissant ses missions. Je me réjouis également de l'adoption de l'amendement visant à prévoir spécifiquement un accès prioritaire à la commission pour les anciens combattants harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local. Il s'agit, là aussi, d'une avancée précieuse pour le travail mémoriel.

1962, la France a reconnu pas à pas, lentement, l'abandon des harkis. De Jacques Chirac à Emmanuel Macron, chaque Président de la République a exprimé la reconnaissance de la Nation envers les harkis et autres supplétifs pour leur engagement aux côtés de la France. Le texte dont nous venons de débattre réaffirme la reconnaissance de la France envers les harkis et vise à réparer financièrement le préjudice subi par les rapatriés ayant transité par un camp ou un hameau. La somme est modeste, reconnaissons-le, et n'est sans doute pas à la hauteur des souffrances subies par les harkis. La distinction entre ceux qui ont été enfermés dans des camps et des hameaux et ceux qui sont venus par eux-mêmes

douloureuse ; encore faudrait-il que la France reconnaisse sa faute, comme l'avait fait Jacques Chirac pour les juifs en 1995. Je voterai ce texte.

Nous avons amélioré le texte, et notre collègue rapporteure, Marie-Pierre Richer, a mené son travail dans un souci d'apaisement. Nous serons donc nombreux à voter ce projet de loi, qui reconnaît la responsabilité de la Nation dans l'abandon des anciens membres des formations supplétives de l'armée française et dans l'indignité des conditions d'accueil, de vie et de séjour au sein de structures privatives de liberté. de l'amendement que notre groupe a soutenu permettra à la commission nationale indépendante de proposer toute mesure de reconnaissance et de réparation pour tous ceux qui ont séjourné dans des structures non couvertes par le texte, afin de prendre en compte toutes les situations dramatiques qu'ont pu connaître les harkis.

simple réparation forfaitaire, sans examen de la situation particulière, c'est-à-dire sans passer par l'histoire individuelle, laquelle a aussi besoin de reconnaissance au-delà de la reconnaissance générale donnée au collectif.

projet de loi portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.